La séance est reprise.

Le mécanisme du plafond mordant permet la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d’action des agences, alors même que le onzième programme élargit leur champ d’action.

Evelyne Corbière Naminzo. Nous sommes nombreux, sur ces travées, à présenter le même amendement, qui reflète notre inquiétude commune quant à la pérennité des moyens alloués aux chambres d’agriculture.

Varenne de l’eau, fourniture d’informations sur la réglementation et les contrôles, réduction de l’usage des produits phytosanitaires, déploiement de la planification écologique, tenue d’un registre des actifs agricoles, déploiement du pacte en faveur de la haie, animation des concertations régionales sur le pacte et la loi d’orientation et d’avenir agricoles. Cette liste, loin d’être exhaustive, reflète l’importance des chambres d’agriculture dans notre pays. Face aux défis qui s’imposent au monde agricole, un accompagnement renforcé, de proximité, en ingénierie et en technicité, est essentiel.

faute d’une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l’inflation. En effet, le montant attribué aux chambres d’agriculture est plafonné et la base cadastrale imposable n’a cessé d’augmenter. Cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux chambres d’agriculture et à l’appauvrissement

au sport de haut niveau. Alors que de nombreuses fédérations sportives se trouvent dans une situation financière dégradée, voire fragile, alors qu’elles font face à la hausse des coûts de l’énergie depuis maintenant près de deux ans et que de nombreuses infrastructures sportives nécessitent des rénovations, je m’interroge. Monsieur le ministre, les

Voilà une occasion unique d’amorcer une réforme structurante de notre service public du sport, et notamment de son financement, en faveur d’une culture sportive pour toutes et pour tous.

35 millions de licenciés en France, qui ont besoin du soutien du Gouvernement et de l’État ! est à M. Thomas Dossus. Cet amendement a pour objet d’augmenter le plafond de deux des taxes affectées à l’ANS : le prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux (FDJ) hors paris sportifs et le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FDJ et des nouveaux opérateurs L’augmentation du plafond de ces deux taxes est d’autant plus justifiée que, depuis plusieurs années, nous constatons une baisse de rendement de la troisième taxe affectée à l’ANS, la taxe Buffet. Les deux plafonds proposés ne sortent pas de nulle part : ils correspondent aux recommandations contenues

que les paris sportifs et les jeux d’argent financent le sport pour une part minoritaire

Coupe du monde de rugby en 2023, jeux Olympiques d’été en 2024, jeux Olympiques d’hiver en 2030 : à quoi cela sert il de financer, de réaliser, de défendre ces grands projets si ce n’est pas pour inciter les Français à faire du sport ?

du Conservatoire, dont le budget actuel repose sur les recettes de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel. La loi de finances pour 2012 a plafonné la ressource affectée à l’établissement à 37 millions d’euros ; ce plafond a déjà été relevé à deux reprises, pour s’établir aujourd’hui à 40 millions d’euros.

est à Mme Guylène Pantel. Cet amendement vise à annuler complètement la baisse des moyens des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) – 30 millions d’euros par rapport à 2023 – et à corriger le montant qui leur est affecté afin de prendre en compte l’inflation.

Je vous remercie,

Les CCI jouent un rôle crucial dans le soutien aux entreprises, dans la formation et dans l’aménagement du territoire. Elles sont également actives dans la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques prioritaires. La réduction de leurs fonds de roulement compromettrait leur capacité à remplir ces missions vitales pour l’économie nationale. En conséquence,

un avis défavorable sur ces amendements.

par l’Autorité nationale des jeux en 2021 révèle que, malgré l’interdiction de la vente de jeux d’argent et de hasard aux mineurs, 34,8 % des jeunes de 15 à 17 ans se déclarent joueurs, 12,1

L’interdiction pure et simple des casinos en ligne revient en effet aujourd’hui à l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux, qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risque. trois Français sur quatre sont favorables à la régulation et au contrôle par l’État des jeux de casino en ligne selon une étude Toluna – Harris Interactive de 2023. Pour remédier à cette situation et protéger les 3 millions de Français qui fréquentent cette offre illégale, nous proposons, par cet amendement, d’encadrer la pratique des casinos en ligne, tout en les assujettissant à un double prélèvement sur le chiffre d’affaires ou produit brut des jeux. Un premier prélèvement serait instauré au profit de l’Agence nationale du sport. Un second second prélèvement serait instauré au profit du budget de l’État et des communes accueillant un établissement de jeux, afin de préserver l’équilibre des filières et de sécuriser ainsi les recettes fiscales des collectivités locales financées par les jeux. Quel

des grands stades de l’Euro 2016, nous proposons, en collaboration avec l’Association nationale des élus en charge du sport, une surtaxe – toujours de 0,3 % – sur les paris sportifs afin de financer les 573 maisons sport santé qui irriguent notre territoire. En effet, l’association alerte

Il faut du temps pour analyser la course et les chevaux. Cette mécanique de jeu est la seule dont dispose le PMU depuis 1891, quand les autres acteurs des jeux d’argent ont pu élargir leur gamme au fil des ans.

par cet amendement, de créer de nouveaux prélèvements au profit de l’État, applicables à une nouvelle offre de loterie hippique qui devrait permettre de renouveler et d’élargir le public du PMU sous le contrôle de l’Autorité nationale des jeux. Cette nouvelle offre de jeux hippiques serait proposée uniquement par le réseau physique de distribution et le PMU serait le seul à pouvoir l’exploiter. Le régime des prélèvements applicables au profit de l’État serait aligné sur le régime existant en matière de jeux de loterie. Cette nouvelle offre de jeux hippiques ne remet en cause ni les équilibres de la Française des jeux ni, plus généralement, ceux des jeux. Elle s’inscrit dans la préservation de l’équilibre des filières voulue par la loi Pacte en 2019.

le taux national de cette taxe à compter de 2024.

J’en reviens au présent amendement. Depuis la suppression de la contribution à l’audiovisuel public quelques semaines seulement après l’élection présidentielle de 2022, plusieurs propositions parlementaires ont émergé pour la remplacer. Jusqu’à présent, ni le Gouvernement ni les majorités parlementaires ne s’en sont emparés.

Ni dépendance politique ni dépendance commerciale : voilà notre ligne. Depuis 2022, nous proposons donc d’instaurer une redevance progressive. L’absence de progressivité de la contribution à l’audiovisuel public était sa principale limite. Nous proposons de créer quatre taux correspondants à quatre tranches de revenus. Cette proposition de l’économiste Julia Cagé est également soutenue par David Assouline. À l’heure actuelle, nous ne savons strictement rien du mode de financement qui sera retenu après 2024. Comme l’écrit le rapporteur pour avis de la commission de la culture, la méthode qui nous est proposée par le Gouvernement n’est pas satisfaisante : ces enjeux méritent un débat d’une autre ampleur pour consolider le service public de l’audiovisuel.